provoquant la condamnation et l'indignation de tous. Ces actes succèdent à des profanations d'édifices catholiques- sept ont été recensées la première semaine de février. Tout se passe comme si, à la crise sociale, à la crise territoriale, s'ajoutait une crise encore plus grave. Plus grave, parce que c'est celle du coeur, qui touche à l'essence même de notre humanité, à l'intimité de chacun de nous, à notre histoire personnelle et collective. La République, parce qu'elle est laïque,

Quelles dispositions comptez-vous prendre pour que chaque citoyen puisse aspirer à une spiritualité apaisée et que la France reste le pays de la liberté, des Lumières et ne devienne pas celui de la barbarie et de l'obscurantisme ? Ne pensez-vous pas que le moment est venu de nommer les fauteurs de troubles ?

vous m'interrogez sur la multiplication des actes antisémites, sur la multiplication des actes de profanation de lieux de culte catholiques ou juifs, sur le climat nauséabond qui se développe dans notre pays. Vous me posez cette question avec beaucoup de gravité, marquant votre indignation et soulignant que vous ne pouvez pas vous contenter de cette indignation. Vous me dites souhaiter qu'en réponse à ces actes

répugnants, qui prennent des formes extrêmement variées : des menaces contre les personnes, des tags, des atteintes contre les symboles. Vous avez vu, comme moi, et je sais que nous aurons l'occasion au cours de cette séance de questions d'évoquer ce sujet, l'atteinte faite à la mémoire d'Ilan Halimi à Sainte-Geneviève-des-Bois. Face à cette multiplication d'actes antisémites ou anticatholiques visant des églises et des cimetières, vous faites bien de rappeler que la République respecte le sacré. sacré. En France, dans notre République, nous avons le droit de croire ou de ne pas croire et, lorsque nous croyons, nous devons être respectés parce que nous croyons. Toujours en France et toujours sous la République, on a respecté les églises, les cimetières, les lieux de culte. Il est impératif de rappeler qu'il doit toujours en être ainsi. Cela ne suffit pas de le dire, j'en ai parfaitement conscience, mais vous savez comme moi que le jour où nous ne le dirions plus, alors, tout serait perdu ! Nous devons donc rappeler la norme, qui est que, en France, on respecte les lieux sacrés, symboles de la République, les lieux de culte, les lieux où reposent les morts.

Nous devons livrer ce combat à l'école, partout, et nous savons qu'il est difficile. Je me souviens, monsieur le président, que l'expression « hussards noirs » désignait autant la couleur revêtus les instituteurs que la logique de combat qui les inspirait : le combat contre l'obscurantisme. Il faut que nous retrouvions, d'une certaine façon, cette logique et que nous livrions absolument partout et en tous lieux ce combat contre l'obscurantisme, contre la haine, contre les préjugés, contre la bêtise la plus crasse, contre la méchanceté la plus vive.

car ce serait trop simple, l'apanage d'une famille politique ; il s'est déployé dans de très nombreuses familles politiques, a imprégné de très nombreux aspects de la société française,

Tous ces éléments, toutes ces constituantes de l'antisémitisme qui se développent dans notre pays doivent être combattus et nommés, avec une indéfectible détermination. Je voudrais assurer le Sénat, que je sais attaché à cette cause, de l'indéfectible détermination de l'ensemble des membres du Gouvernement sur ce sujet. La parole est à M. Dominique de Dominique de Legge, pour la réplique. Merci, monsieur le Premier ministre, de cette réponse, mais je crois, et vous l'avez souligné, qu'il faut avoir le courage de nommer les auteurs. Les auteurs, on les connaît, c'est l'extrême gauche antisioniste, c'est l'islam radical qui veut imposer la charia, c'est le nazisme et c'est l'extrême droite, qui regrette cette période de la France. Alors, permettez-moi de vous inviter très respectueusement à méditer cette belle phrase d'Albert Camus

Révulsés et affligés, nous affichons notre solidarité à l'égard de la communauté juive et nous condamnons avec force les insupportables profanations de tous les lieux de culte qui se multiplient dans les églises, synagogues et mosquées. Cela doit cesser Sans faire d'amalgame, il n'échappe à personne que le mouvement des « gilets jaunes » est aussi générateur d'appels à la haine. Chaque samedi, ces défilés entretiennent en France un climat nauséabond fait de populisme et d'antiparlementarisme. Pourtant, il ne s'agit plus que d'une poignée de Français, dont une partie d'extrémistes, et qui ne représentent qu'eux-mêmes ! Dans une démocratie, les représentants doivent être élus, dois-je le rappeler ici ? Vous recevez comme moi, chers collègues, des courriers insensés qui nous appellent, entre autres choses, à la destitution du Président Macron. Au diable l'État de droit et le résultat des élections Peu importent aussi les conséquences économiques et les salariés mis au chômage technique ! Vous n'êtes pas sans savoir, monsieur le ministre, que les commerçants expriment de plus en plus fort leur ras-le-bol, quand ils ne descendent pas, eux aussi, dans la rue, comme à Toulouse. Cette exaspération gagne désormais les élus municipaux, qui sollicitent le Gouvernement auquel ils demandent une indemnisation pour les villes touchées par les dégradations à l'issue des manifestations. L'agitation de rue doit cesser ! S'ils veulent manifester, très bien, mais selon les règles républicaines : pas n'importe où, pas n'importe comment Le mandat d'Emmanuel Macron s'achèvera dans 166 semaines. Au train où vont les choses, peut-on imaginer qu'il y aura un acte LCXVI des « gilets jaunes » ? Monsieur le ministre, ma question est simple : quand comptez-vous faire rétablir l'ordre républicain ?

Réforme longtemps annoncée, demandée et attendue par les contribuables mais jamais mise en oeuvre, le prélèvement à la source est aujourd'hui soutenu par les trois quarts des Françaises et des Français.

Le pari que les entreprises françaises s'organiseraient en temps et en heure pour que ce prélèvement soit effectif et bien compris sur les fiches de paye de leurs salariés, mentionnant, par exemple, à titre d'information sur les dernières fiches de paye 2018 quel serait le salaire versé après le prélèvement à la source. Le pari que les cinq millions de foyers bénéficiant d'un crédit d'impôt pour service à la personne ou pour frais de garde d'enfant percevraient ce crédit d'impôt sous forme d'avance de 60 % versée dès le 15 janvier et correspondant au crédit ou à la réduction d'impôt de l'année précédente, avant le versement de la totalité à l'été 2019. Enfin, le pari que votre ministère et les fonctionnaires de votre administration déploieraient, pendant plusieurs mois et le temps nécessaire, des moyens de communication, d'information et d'accompagnement à la hauteur de cet enjeu. Ce succès montre la préparation de la réforme. Avant l'été dernier, un sondage montrait que les deux tiers des Français payant l'impôt sur le revenu se sentaient bien informés. Ce succès montre aussi que les Cassandre en tout genre, prompts à souhaiter l'échec du Gouvernement plutôt que la réussite collective, se sont trompés. gaz. C'est une usine à gaz ! Une proposition de loi pour retarder encore la réforme a même été déposée. Votre question ! Alors, monsieur le secrétaire d'État, si la mise en oeuvre du prélèvement à la source est d'ores et déjà un succès, ce succès, nous le devons à la fois aux entreprises et collecteurs. Il faut maintenant transformer définitivement l'essai. Pouvez-vous nous expliquer les mesures qui sont prises pour assurer, durant cette année 2019, l'accompagnement des entreprises ? Quels sont les moyens ... Terminez ! ... mis en oeuvre dans votre administration pour répondre aux questions

Il n'y a eu aucun systémique et l'ensemble des contribuables paient désormais un impôt contemporain, ce qui est l'objectif principal. En effet, 7 millions de contribuables français voient leurs revenus varier

Lundi 11 février, les arbres plantés à Sainte-Geneviève-des-Bois à la mémoire d'Ilan Halimi ont été coupés, profanés. J'étais maire de cette commune en 2006 quand Ilan a été retrouvé agonisant, le long de cette voie ferrée, après vingt-quatre jours de terribles tortures. Enlevé, frappé, brûlé, torturé, Ilan est mort simplement parce qu'il était juif. Personne ne pouvait plus ignorer qu'on pouvait de nouveau s'en prendre à un juif en France en pensant s'en prendre à une famille, à une communauté privilégiée, qui n'aurait aucun mal à payer une forte somme d'argent pour obtenir sa libération. L'assassinat d'Ilan avait malheureusement un caractère annonciateur. Car, il faut le dire, depuis ce 13 février 2006, mourir en France parce qu'on est juif n'est malheureusement plus si exceptionnel que cela. Il faut le dire aussi, les condamnations de principe ne sont plus suffisantes, les cérémonies commémoratives et les minutes de silence ne peuvent plus être les seules réponses à l'intolérable. Alors, je sais que vous allez me dire, à raison, que beaucoup de choses sont initiées pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme. J'étais d'ailleurs avec vous, monsieur le Premier ministre, à Matignon, mardi, pour la remise du prix Ilan Halimi à des jeunes engagés contre ce fléau. Je sais que vous allez me dire, à raison, que des actions sont engagées pour la formation des personnels, des enseignants, des policiers, des magistrats. Je sais que vous allez me dire, à raison, qu'il faut adapter la loi pour agir plus sévèrement face aux messages haineux sur les réseaux sociaux. Mais, monsieur le Premier ministre, ne pensez-vous pas que l'enjeu de la fraternité dans notre pays mérite une action encore plus résolue, des actions encore plus rapides et encore plus fortes ? Nous savons le rôle de l'éducation pour répondre à ce défi et nous savons aussi qu'aujourd'hui, en 2019, des projets pédagogiques, associatifs ou institutionnels auprès de la jeunesse ne sont pas menés, faute de moyens. Ne pensez-vous pas que la gravité de la situation impose que notre pays consacre plus que 6 millions d'euros par an à la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT,

J'ai eu l'occasion de le dire- vous vous en souvenez peut-être -face à tous ces coups terribles que nous prenons, face à tous ces actes antisémites, face non pas au découragement

Oui, il faut former ! Oui, il faut éduquer ! Oui, il faut dénoncer ! Oui, il ne faut jamais renoncer ! Mais c'est un combat long, je le sais. Les phrases que je prononce ont été dites avant moi, peut-être avec plus de talent mais pas avec moins de détermination, par des Premiers ministres qui se sont pleinement engagés dans la lutte contre l'antisémitisme.

que le Gouvernement travaillait sur des mesures qui permettraient de ne pas avoir de hausse. Il nous disait même : « Dans un mois, les tarifs de l'énergie vont baisser, je peux le garantir aux Français, de 2 % à 3 %. » %. » Aujourd'hui, c'est une hausse de 6 % des tarifs qui est annoncée, la hausse pouvant même être plus importante pour le mois de juin. Après la mobilité, vous allez créer de nouvelles fractures territoriales vous prenez le risque de faire basculer dans la précarité énergétique de nouveaux ménages, alors qu'ils sont déjà près de 6 millions dans notre pays ! Vous demandez encore une fois à nos concitoyens de payer plus. Vous leur demandez de payer, alors que ces hausses successives ne sont que le reflet de l'échec de la libéralisation du marché de l'électricité. Vous leur demandez de se résoudre à accepter une répercussion sur leurs factures de plus de 100 euros par an, alors que toutes les demandes de revalorisation du SMIC, de véritable négociation sur les salaires sont balayées d'un revers de main en ce moment même. Hausse des prix du carburant, hausse des prix alimentaires, hausse des prix de l'énergie, gaz et électricité : c'est une véritable politique assumée de paupérisation de nos concitoyens que vous menez actuellement. Monsieur le ministre, quelles dispositions pérennes allez-vous prendre pour endiguer ce phénomène continu d'augmentation artificielle du prix de l'électricité ? Quand accepterez-vous de baisser les taxes sur ce bien de première nécessité ? CTA, TFCE, TVA, CSPE : autant de taxes qui pèsent pour près d'un tiers dans la facture des ménages de notre pays ! Vous l'avez fait pour ADP et pour les dans le cadre de la préparation du Brexit, pourquoi ne pas le faire, une bonne fois pour toutes, au profit de nos concitoyens ? La parole

cette année, alors, vous le savez très bien, cela serait répercuté encore plus fort l'année prochaine. Nous avons pris un engagement : pas de hausse des tarifs de l'électricité pendant l'hiver. Nous tenons cet engagement pour que cette hausse ne s'applique pas pendant les périodes où nos compatriotes se chauffent.

l'hiver sera quand même rude, et l'augmentation de cet été sera répercutée sur les factures de nos concitoyens l'hiver prochain. Vous ne réglez pas la question du pouvoir d'achat dans notre pays

croix gammées sur les portraits de Simone Veil, « » badigeonné sur la devanture d'un restaurant, arbres plantés en hommage à Ilan Halimi, ce jeune homme enlevé, séquestré et torturé à mort parce qu'il était juif, sciés l'hydre toujours renaît ! Ces actes, d'une singulière lâcheté, révèlent un antisémitisme qui ne s'estompe pas, qui reste, qui mute ; un antisémitisme qui porte atteinte à la communauté nationale, qui percute nos valeurs républicaines, qui questionne notre devoir de mémoire ; un antisémitisme désinhibé par internet et les réseaux sociaux, sur lesquels prospèrent les mythes complotistes, des slogans tout droit sortis des poubelles de l'histoire, une insondable passion pour la haine. Les actes et les menaces antisémites ont crû de 74 % l'an dernier. Ils traduisent une réalité vécue et ressentie tous les jours par de nombreux Français qui subissent des injures, des violences, en raison de leur kippa ou de leur patronyme, dans la rue, dans les transports, sur internet, à l'école ou devant leur lieu de culte. Nous ne pouvons accepter que nos compatriotes de religion ou de culture juives ne puissent vivre en sécurité simplement du fait de ce qu'ils sont. À ceux qui se croient imperméables, rappelons les mots de Frantz Fanon : « Quand vous entendez dire du mal des juifs, dressez l'oreille, on parle de vous. Monsieur le Premier ministre, quelles mesures le Gouvernement entend-il prendre pour lutter contre cet antisémitisme qui sème la honte et l'horreur dans la République, au pays des droits de l'homme ? Cette lutte nécessite l'engagement de toutes et de tous, et nous serons aux côtés de toutes celles et de tous ceux qui s'y engageront. La parole

qui nous permet de les détecter et de demander aux fournisseurs d'accès à internet de procéder à des retraits. Nous procédons également à de longues investigations judiciaires qui nous permettent de confondre leurs auteurs ; de ce fait, de nombreuses condamnations

sécuriser physiquement les cérémonies, les lieux de manifestation et les fêtes les plus importants. Nous menons là encore cette action de manière extrêmement résolue et déterminée ; l'ensemble des fonctionnaires de police et de gendarmerie

Si je la pose officiellement, c'est parce qu'elle est, me semble-t-il, révélatrice d'un malaise. À tort ou à raison, la psychologie collective française veut condamner la classe politique, réduite à son impuissance. son impuissance. Emmanuel Macron a lancé des pistes de réflexion sur les réformes constitutionnelles. Je veux rebondir sur l'une d'entre elles : l'amélioration de la qualité de la loi.

Certes, nous sommes réticents lorsqu'il s'agit de toucher à nos droits parlementaires. Néanmoins, à l'instar d'autres pays, le Sénat a déjà expérimenté des procédures d'adoption simplifiées. Tancés pour notre lenteur, permettez-nous, monsieur le ministre, à notre tour, de vous tancer sur la vôtre, celle de l'exécutif.

Des décrets d'application sont prévus, après avis de la CNIL et du Conseil d'État. Nous sommes le 14 février 2019 ! Déjà sept mois d'attente, et les caméras sont toujours sagement rangées dans les tiroirs Monsieur le ministre, par votre action, ce dispositif des caméras-piétons a démontré son efficacité. À l'heure où les violences s'inscrivent désormais dans le rituel du samedi, pourriez-vous réfléchir également à accélérer le temps réglementaire ? Je ne mets pas en cause la qualité du travail fourni par vos services, mais je veux dénoncer ce décalage, incompris par l'opinion publique, entre la décision politique et sa concrétisation.

de police municipale, tout comme nous protégeons les fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales dans l'utilisation de ce dispositif. Je peux en tout cas vous assurer qu'il n'y a aucune volonté du Gouvernement de ne pas mettre en oeuvre ces dispositions.

Bien évidemment, tout le monde s'inquiète pour 2019, car il n'y a aucune chance que la situation s'améliore. Cela pénalise évidemment les Français qui attendent un logement social, mais cela pénalisera aussi les communes, auxquelles, au titre de l'article 55 de la loi SRU, on assigne des objectifs de construction de logements sociaux. En 2015, le CGEDD, organisme d'État, avait déjà tiré la sonnette d'alarme en nous prévenant que les deux tiers des communes risquaient d'être carencées en 2019, parce que les objectifs assignés étaient trop importants. l'on y ajoute la crise du logement social, que vous avez créée par vos choix politiques, vous allez mettre beaucoup de communes dans une très grande difficulté ! Alors, monsieur le ministre, quelles instructions le Gouvernement entend-il donner aux préfets de région, qui président les comités régionaux de l'habitat, pour que cette difficulté soit prise en compte au moment où sera jugée la bonne volonté des maires pour la construction de logement social ? La

ministre, au moins sur le constat, nous devrions pouvoir tomber d'accord : il y a urgence pour le logement social ! Ici, au Sénat, des Républicains au parti communiste, à l'automne 2017 comme à l'automne 2018, tout le monde vous a dit que vos décisions allaient précipiter le secteur dans une crise.

Union Centriste. Madame la ministre des solidarités et de la santé, l'épidémie de grippe touche de plein fouet notre pays ; elle est à son niveau maximum. Depuis le mois de janvier, nous dénombrons, hélas, près de 1 100 décès 1 100 décès ! Nos services d'urgence ne désemplissent pas. Les complications respiratoires, ainsi que l'embouteillage classique des salles d'attente, expliquent en partie ce phénomène. Dans le département de l'Essonne, à l'hôpital d'Arpajon, un médecin réanimateur expliquait à France 3 que la priorité était donnée aux urgences virales. Il indiquait que huit lits supplémentaires avaient été ouverts cette année. Surtout, des interventions programmées et des prises en charge de chimiothérapies ont dû être décalées. C'est donc un sujet de santé publique sérieux, qui n'est pas à prendre à la légère. Ce sujet concerne l'ensemble des Français. Parmi la population, les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans et les enfants sont les plus touchés, car ils sont les plus fragiles. Selon l'Agence nationale de santé publique, les résultats préliminaires disponibles en semaine 5 indiquent une efficacité vaccinale chez l'ensemble des personnes à risque de 59 % contre le virus A-H1N1 et de 19 % contre le virus A-H3N2. Dans le même temps, toujours selon le bulletin d'information de l'ANSP, la couverture vaccinale en France métropolitaine a progressé de 1,6 % par rapport à l'année dernière pour l'ensemble des sujets à risque. Par conséquent, madame la ministre, plusieurs questions se posent. D'abord, pouvez-vous nous confirmer ce bilan ? Ensuite, même s'il est encore tôt pour tirer des conclusions, qu'en est-il vraiment de l'efficacité du vaccin ? Faudrait-il envisager, comme certains le proposent, une obligation vaccinale pour les publics fragiles et les professionnels exposés ? Enfin, ne conviendrait-il pas de renforcer les campagnes de vaccination et de sensibilisation contre la transmission du virus ? La parole

Ce virus a des conséquences potentiellement graves, surtout pour les sujets fragiles, les personnes âgées et celles qui ont déjà des pathologies chroniques ; cela peut évidemment entraîner le décès

les personnes obèses et les femmes enceintes. Nous avons également le souhait d'augmenter la couverture vaccinale des professionnels soignants ; cette couverture est insuffisante dans nos établissements de santé et nos établissements médico-sociaux. À cette fin, j'ai j'ai pris deux mesures particulières cette année. D'une part, j'ai élargi la possibilité de vaccination dans les pharmacies, en autorisant notamment les primo-vaccinations, ce qui n'était pas le cas auparavant, dans quatre régions françaises. Cela a abouti à 700 000 vaccinations en pharmacie. Cette mesure sera étendue à l'ensemble de la France

Dans le respect de ses valeurs et ses principes, me semble-t-il, vous présentiez hier soir une transformation de la fonction publique aux partenaires sociaux. Nous savons une telle transformation nécessaire, parce que le secteur public, au même titre que le secteur privé, est confronté à des mutations majeures la montée en puissance du digital, notamment de l'intelligence artificielle, mais aussi, dans ce contexte, les exigences nouvelles des usagers pour un meilleur service public. Elle est nécessaire aussi, parce que la fonction publique fait face à un enjeu d'attractivité en raison des attentes des jeunes générations et du manque de mobilité,

Depuis quarante ans, il est demandé aux agents publics de s'adapter, mais on ne leur en donne pas les moyens. Je pense notamment à la formation. Des métiers sont interrogés, remis en cause. Les agents doivent pouvoir bénéficier d'une deuxième carrière, voire d'une troisième, et ne pas être laissés sur le bord de la route. Alors, je comprends que vous proposez, notamment, plus d'autonomie pour les cadres, la reconnaissance du mérite, tant pour les fonctionnaires que pour les contractuels, davantage de mobilité, ainsi que l'égalité de traitement et de carrière entre les hommes et les femmes. Il n'est Il n'est pas envisageable de maintenir un. Quelques syndicats ont pourtant exprimé des réserves. Alors, monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous indiquer la place que vous comptez donner, dans les semaines à venir, aux syndicats, aux associations représentatives des collectivités, au débat parlementaire, en particulier au Sénat, et bien évidemment aux agents publics ?

restant fidèle à ses principes et à ses valeurs, de répondre à la nécessité impérieuse de transformer ce statut, d'apporter des souplesses pour permettre à l'administration d'être plus efficace, mais aussi de donner des droits nouveaux tant aux agents titulaires qu'aux agents contractuels. Nous allons travailler, comme nous l'avons fait depuis un an, avec les organisations syndicales et les employeurs publics, pour mettre en place un dialogue social à la fois plus simplifié, recentré sur l'essentiel et protecteur, pour créer de nouveaux leviers managériaux en matière de diversification des recrutements et d'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels, mais aussi pour mieux tenir compte de l'engagement et du mérite. Nous allons aussi travailler, à l'évidence, sur la question de la formation et des mobilités. C'est sur ce point que vous avez particulièrement insisté, en soulignant combien les employeurs publics doivent être exemplaires en la matière ; nous ne le sommes pas aujourd'hui. C'est le démembrement ! Nous devons permettre à des agents dont le métier est remis en cause par des évolutions technologiques, par des restructurations, par des réorganisations ou par des révisions de politiques publiques de connaître une deuxième ou une troisième carrière. Cela nécessite d'améliorer le système de formation initiale, mais aussi continue des agents. C'est l'occasion pour moi de saluer le travail que vous avez mené avec le député Jacques Savatier Savatier sur le système de formation continue des agents de la fonction publique territoriale. Vous avez remis, mardi dernier, un rapport à M. le Premier ministre sur ce sujet. Ce rapport utile et précieux, parce qu'il explore différents scénarios, est né d'une concertation et de rencontres nombreuses sur le territoire ; il nous permettra de nourrir les travaux en la matière. Vous me demandez quelle place est donnée dans le processus de concertation aux organisations syndicales, aux employeurs et aux parlementaires, ainsi qu'à l'ensemble des agents du service public. Il s'agit d'une place forte : nous avons ouvert une concertation avec les instances représentatives, et j'attends des organisations syndicales des propositions de représentation. Elles n'en veulent pas ! Concernant les parlementaires, votre rapport est l'illustration est l'illustration des enrichissements que le débat parlementaire nous permettra d'apporter à ce texte pour construire une fonction publique moderne, rénovée, protectrice des agents et au service des usagers.

Dans la guerre contre Daech, ce sont les Kurdes qui ont neutralisé plus de 30 000 djihadistes et chassé cette organisation terroriste de tous les territoires qu'elle occupait. Ils ont, pour ce faire, sacrifié des milliers de combattants et se sont révélés être des alliés remarquables. Alors, comment accepter qu'à l'heure de la victoire militaire les Kurdes soient abandonnés par la coalition internationale ? Après le retrait annoncé de l'armée américaine, une fois privés de défense aérienne et d'armes lourdes, les Kurdes, mais aussi leurs alliés arabes et chrétiens, se retrouveront seuls face à une prévisible agression du Président turc et de ses supplétifs islamistes. Nous ne pouvons pas l'accepter d'Afrine, il y a tout juste un an, a déjà entraîné des crimes, des destructions et des déplacements de la population kurde qui s'apparentent à un véritable nettoyage ethnique. Face à une situation très inquiétante, il est indispensable que la France et l'Europe s'engagent aujourd'hui avec force. Des voix s'élèvent pour appeler à une initiative européenne soutenant la création par l'ONU d'une zone de protection dans le nord de la Syrie. Cette zone de protection dissuaderait toute invasion de l'armée turque, ainsi que le retour des troupes du régime syrien. Elle empêcherait l'expansion de l'influence russe et iranienne. Enfin, elle favoriserait une meilleure protection des minorités dans les négociations sur l'avenir de la Syrie. La France a là une occasion historique de sauver l'honneur de la coalition contre Daech en se mobilisant réellement avec ses alliés européens. Pouvons-nous compter sur le Président de la République et sur le Gouvernement pour agir en ce sens ? La

vous l'avez rappelé, nous sommes à la veille d'une étape décisive au Levant. L'engagement militaire de la communauté internationale dans la région vise à défaire Daech et à permettre aux forces irakiennes de contenir sa résurgence. L'opération Chammal, en formant les forces irakiennes et en appuyant les Kurdes syriens et leurs partenaires, permet d'achever la reconquête de l'ultime bastion de Daech. je le dis aujourd'hui, les terroristes s'accrochent aux quelques enclaves qu'il leur reste ou se dissimulent au milieu des populations civiles. ont annoncé leur retrait. Néanmoins, à la suite de discussions, ils ont conditionné ce retrait à la défaite du califat territorial. Il est également essentiel que ce désengagement de Syrie ne soit pas précipité,

part. Nous poursuivons donc nos discussions avec les Américains, au sein de la coalition, pour donner des garanties aux Kurdes de Syrie, contrer les ambitions iraniennes et éviter la dispersion des combattants étrangers. Bien sûr, nous continuerons d'apporter notre soutien aux efforts menés en faveur de la stabilité de la région. Nous ne pouvons abandonner les forces arabes et kurdes, qui ont combattu vaillamment. Une solution négociée sera nécessaire ; elle devra préserver leur sécurité, mais aussi répondre aux préoccupations de sécurité légitimes de la Turquie. qu'il est très complexe, nous restons naturellement attachés à ce qu'une solution politique puisse être apportée globalement à la crise syrienne et nous poursuivrons les échanges avec nos partenaires.

Concertation, discussion, négociation, ouverture, écoute sont les mots que le chef de l'État martèle, à juste titre, dans ses échanges avec les maires et les Français depuis quelques semaines. Il les place haut ! Il en fait l'alpha et l'oméga de sa nouvelle méthode de gouvernance, et il a sans doute raison. Qu'importe que sa conversion au dialogue soit tardive. Elle seule permettra de sortir de la crise, car on ne peut pas réformer la société par voie d'autorité. Cette nouvelle méthode aurait-elle échappé à votre gouvernement, Une réforme de la justice contre l'ensemble des professionnels du droit- magistrats, avocats, greffiers -, sans écouter les propositions du Sénat, qui vous a pourtant tendu la main en organisant une table ronde un projet de loi Santé contre les professionnels du secteur, qui dénoncent tous un texte élaboré sans concertation et dont l'essentiel des propositions sera formalisé par ordonnances ; annonce d'une réduction des dessertes de TGV- je ne crois pas avoir entendu les Français formuler une telle demande, pas même dans les grands débats une carte pénitentiaire imposée aux élus locaux, sans dialogue ni concertation ; des ordonnances pour réformer la politique des déchets ... Dois-je rappeler, ici, le travail colossal des parlementaires sur ce sujet, comme sur d'autres sujets que je viens d'évoquer ? Pourquoi les mettre à distance ? Monsieur le Premier ministre, comme vous pouvez le constater, les exemples ne manquent pas. Ils sont nombreux. Je suis pourtant convaincu que la voie de l'apaisement est celle que vous recherchez. Alors, qu'attendez-vous pour mettre en oeuvre dans votre politique la seule méthode qui vaille, celle de la concertation ?

Le Président de la République et le Premier ministre ont annoncé un certain nombre d'étapes qui, nécessairement, auront leur traduction législative. La discussion aura alors lieu au Parlement. Nous comptons bien que celui-ci puisse se saisir de ces questions,

Républicains. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Elle porte sur l'avenir que vous avez le pouvoir de réserver aux 240 salariés de l'entreprise Arjowiggins Security, dont la liquidation judiciaire a été brutalement annoncée à la mi-janvier,

Arjowiggins est le coeur battant de tout un territoire en Seine-et-Marne, le nôtre ! Elle dispose d'un savoir-faire exceptionnel pour fabriquer le papier sécurisé français pour nos passeports, cartes d'identité, cartes grises, permis de conduire. Aujourd'hui, la seule en France ! À ce jour, nous en sommes réduits à mendier auprès de la ministre du travail pour obtenir un PSE digne pour les salariés. Je suis sénatrice de Seine-et-Marne, et je veux faire part à la Haute Assemblée de mon indignation face à votre mutisme. J'ai écrit au Président de la République pour l'alerter sur l'extrême urgence à intervenir. Pas de réponse ! Je vous ai adressé une copie de ce courrier, ainsi qu'à Bruno Le Maire. Pas de réponse ! Hier, Christian Jacob vous a posé une question. Pas de réaction, ou si peu ! Que faut-il faire pour attirer votre attention ? Il serait inconcevable que la France ne fabrique pas elle-même son papier sécurisé pour ses documents officiels. C'est en France qu'il faut le faire, et pas ailleurs Qui d'autre qu'Arjowiggins pour le faire ? C'est une question, non seulement d'ambition, de stratégie, mais aussi de sécurité nationale. Qu'attendez-vous, monsieur le Premier ministre, pour mobiliser un financement en vue d'aider ces salariés remarquables, investis et responsables, à créer une société coopérative et participative ? Qu'attendez-vous pour vous déplacer sur le terrain ? Les salariés se désespèrent d'obtenir votre aide concrète, et nous aussi des comptes publics. Madame la sénatrice, vous appelez l'attention du Gouvernement sur la situation de la société Arjowiggins Security de Jouy-sur-Morin, qui a été placée, comme l'ensemble des sociétés du groupe Arjowiggins, en liquidation judiciaire le 30 janvier dernier.

Dans ce cadre, le repreneur s'était engagé devant le tribunal à limiter les suppressions d'emplois et à soutenir cette société dans ses efforts de modernisation et de recherche de nouveaux marchés. Il s'était également engagé à subvenir au financement des opérations par le biais de divers instruments bancaires, notamment l'obtention de garanties d'un montant de 7 Quelques mois à peine après la reprise, le groupe BMT n'avait proposé aucun plan industriel crédible et a toujours refusé d'octroyer le moindre euro pour remédier à une situation financière très dégradée. rappelés -, y compris sur le plan financier, et l'attitude constructive des salariés, qu'il faut saluer, car ils se sont montrés systématiquement ouverts pour améliorer la compétitivité du site, la déclaration de liquidation judiciaire confirme l'échec du groupe BMT et l'irresponsabilité

engagement total de l'État pour trouver des solutions, mais il a aussi souligné devant l'Assemblée nationale, comme je me permets de le faire devant le Sénat, le caractère extrêmement dégradé de la situation. Vous connaissez ce site, madame la sénatrice, et sa situation financière. Nous pouvons ensemble dénoncer l'irresponsabilité de tel ou tel acteur économique privé ne tenant pas les engagements qu'il a pris et les risques qu'un tel comportement fait peser sur ce secteur. Il faut regarder cette réalité en face et travailler de concert. La question posée, hier, par le président Jacob augurait d'une vraie capacité des élus à se rassembler, avec le Gouvernement, pour chercher ensemble toutes les solutions possibles.

relative au délai d'intervention du juge des libertés et de la détention en rétention administrative à Mayotte. Dans la suite de

La séance est reprise. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative au délai d'intervention du juge des libertés et de la détention

Cette dérogation au droit commun avait effectivement été supprimée par erreur dans la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie.

nous ne pouvons adopter cette proposition de loi au seul motif qu'elle vient corriger une erreur sans examiner au préalable la pertinence du dispositif qu'elle entend rétablir. Pour mémoire, le délai de cinq jours avait été introduit à l'article 31 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique,

avait pour objet de garantir, dans le contexte migratoire particulier qui y prévaut, la mise en oeuvre effective à Mayotte des principes des réformes contentieuses de la loi du 7 mars 2016. Ayant lu avec attention le rapport il en ressort effectivement et très nettement que la pression migratoire sur son territoire est extrêmement forte- affolante, même. Ainsi, 48 % de la population de Mayotte est de nationalité étrangère, soit 120 000 personnes pour une population d'environ 256 000 Les estimations du nombre d'étrangers en situation irrégulière oscillent entre 60 000 et 75 000 personnes, chiffres très probablement sous-estimés. Nous pouvons aisément imaginer le grand nombre de dossiers que le territoire doit traiter. Les représentants de la préfecture, lors de leur audition, ont ainsi fait part de leurs craintes quant aux conséquences difficilement surmontables d'une réduction du délai à deux jours. Le délai dérogatoire de cinq jours fait donc largement consensus, tant pour le Gouvernement que pour la majorité des groupes parlementaires. Aussi, le groupe du RDSE votera à l'unanimité en faveur de cette proposition de loi. Je veux néanmoins rappeler, à toutes fins utiles, que, lors de l'examen de la loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie par la Haute Assemblée en juin 2018,

; la difficile question des mineurs, même accompagnés ; la nécessaire réflexion sur le codéveloppement partout où les États vacillent et où il y a de la détresse économique économique ; l'impérieuse nécessité, enfin, de confier un rôle plus important aux élus locaux dans la procédure des régularisations administratives. À titre d'illustration sur ce dernier point, j'avais suggéré la création d'un office des migrations à Saint-Martin, pour mieux coordonner délivrance des titres de séjours et délivrance

Pour l'heure, au vu des délais contraints, le groupe du RDSE suivra les auteurs de la proposition de loi, afin que celle-ci soit adoptée avant le 1 mars 2019, raison pour laquelle nous n'avons pas proposé d'amendements. Mayotte, au regard de la pression migratoire exceptionnelle qui s'exerce sur son territoire, mérite que lui soit appliquée une législation différenciée. secrétaire d'État, mes chers collègues, cela ne réglera pas ce problème, beaucoup plus profond et dont il faudra bien, un jour, se saisir.

». Or, on le voit bien, du fait de la rigidité de nos systèmes d'organisation, du fait des garanties qu'il faut prendre pour renforcer les services avec des personnels qualifiés, dans un certain nombre de situations qui engagent l'application du droit sur des questions qui ne sont pas mineures, on est bien obligé de trouver des dispositifs d'adaptation, sans simplement se réfugier derrière l'augmentation indéfinie des moyens. C'est

Le droit du sol n'est pas supprimé à Mayotte ! Que vous continuiez à ne pas être d'accord avec les dispositions qui ont été votées et qu'Alain Richard vient de rappeler, nonobstant les décisions du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel, c'est votre droit le plus absolu,

Il organise les audiences, prenant en compte la situation très particulière de Mayotte, en conservant une égalité sur la durée totale de rétention, qui reste de quarante-cinq jours au maximum. L'article revient au droit existant avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 mars. C'est justifié par les contraintes pratiques que subit le juge des libertés et de la détention et par le nombre très élevé de contentieux. » Ces propos sont ceux d'Ericka Bareigts, alors ministre des outre-mer, qui défendait cet amendement

est ainsi libellé : La parole est à M. Xavier Iacovelli. Cet amendement a pour objet d'interdire en toute hypothèse le placement en rétention d'un mineur, qu'il s'agisse d'un mineur accompagné ou d'un mineur isolé, l'intérêt supérieur de l'enfant ne devant souffrir aucune exception. Cette interdiction est d'autant plus urgente que, à Mayotte, ce sont près de 4 000 mineurs qui sont retenus chaque année en centre de rétention administrative. En vertu de cette proposition de loi, ces enfants pourraient désormais être retenus sans pouvoir saisir le juge des libertés et de la détention avant le sixième jour et, ce faisant, faire l'objet d'un éloignement sans que le juge ait été saisi et ait pu statuer sur la légalité et la régularité de leur rétention. Quel

Ce sujet est beaucoup trop sérieux pour que nous l'abordions ainsi au détour d'une proposition de loi technique sur Mayotte. En tout état de cause, un amendement identique a déjà été rejeté par la commission des lois, puis par le Sénat, lors de l'examen de la loi Immigration, asile, intégration. La position du rapporteur à l'époque, notre collègue François-Noël Buffet, avait été de limiter, mais non pas d'interdire, la rétention des mineurs. Par cohérence, je vous propose de réserver le même sort à cet amendement et de le rejeter. L'avis est donc défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement ?

de la préfecture de Mayotte nous avaient dit eux-mêmes qu'ils allaient un peu au-delà de ce qui était prévu par les textes.

L'objet de cette proposition de loi est de réparer un défaut de coordination dans la rédaction d'un texte à l'Assemblée nationale. Je ne reviendrai pas sur la nécessité de rétablir à Mayotte un délai de rétention administrative de cinq jours

Je voudrais simplement ajouter que cette correction ne saurait devenir le prétexte à une surenchère démagogique, d'un bord ou d'un autre. La situation à Mayotte, vous l'avez compris, chers collègues, est très difficile.

de l'État voisin, qui revendique ouvertement la souveraineté sur Mayotte. Les Mahorais ont sans cesse à coeur la volonté d'être reconnus comme Français à part entière- cela remonte à loin -et la crainte de ne pouvoir vivre décemment et éduquer leurs enfants correctement, compte tenu de l'insuffisance énorme des infrastructures, de la pauvreté et de l'insécurité qui règne. Aussi, toute disposition relative aux étrangers doit être étudiée avec la plus extrême attention, dans le respect de la population mahoraise, qui vit au quotidien des difficultés dont on ne mesure pas l'ampleur dans l'Hexagone, sauf peut-être quand les troubles sociaux paralysent l'île plusieurs mois. ce n'est pas que les Mahorais ne sont pas respectueux des droits de tout être humain : leurs traditions d'accueil tout au long de leur histoire peuvent en témoigner. Mais comment faire face aux milliers d'arrivées chaque année, alors que 84 % de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté, que les enfants vont par rotation à l'école et que les bidonvilles s'étalent sur des collines inconstructibles Abordons donc les amendements qui nous sont proposés- et dont plusieurs ont été déclarés irrecevables -avec la plus grande prudence. D'ailleurs, une mesure qui semble séduisante peut engendrer de redoutables effets pervers. Pas de précipitation donc, même si cette proposition de loi de simple coordination légistique n'est sans doute pas le véhicule le plus approprié pour tenter de répondre à l'ensemble des inquiétudes et des attentes des Mahorais.

ne nions pas, bien entendu, que le département de Mayotte fait face à une situation dramatique, avec une pression migratoire qu'aucun autre département français ne connaît.

le partage ici. Une action diplomatique auprès des Comores, la lutte contre l'immigration irrégulière et contre les passeurs, une politique économique et sociale globale, qui incorpore aussi la situation comorienne : voilà la solution durable à cette situation En revanche, il est absolument impossible d'imaginer que c'est un recul des droits et des libertés fondamentales qui serait une réponse adaptée : on ne peut prétendre cela ni dans l'Hexagone ni à Mayotte.

des Mahorais- des avocats, des associations -constatent sur le terrain que la pente dangereuse sur laquelle le territoire de Mayotte s'engage avec la France n'est pas une solution.

J'en avais déposé cinq, issus d'ailleurs des réflexions de notre ami Mansour Kamardine, mais quatre d'entre eux ont été déclarés irrecevables. Je me vois donc complètement désarmé par l'article 45

Un tel débat de fond, qui est pertinent, mériterait d'avoir lieu à l'occasion de l'examen d'un texte de loi spécifique, et non au détour de cette proposition de loi technique destinée à corriger une erreur de coordination. Adopter cet amendement, c'est prendre le risque de manquer la date butoir du 1 mars et de relancer la navette. Je rappelle que, faute d'un vote de ce texte dans les mêmes termes

Elle semble même aller à l'inverse de la volonté de son auteur. En effet, l'amendement vise des troubles à l'ordre public dans des cas où, actuellement, une simple menace suffit.

vous avez naturellement été sensible, et vous l'êtes encore, à la nécessité que la loi garde sa cohésion et ne soit pas déformée par la dispersion des articles qui la rendent parfois obèse en abordant de multiples sujets.

que je suis d'accord avec vous. Nous avons eu hier après-midi un débat provoqué par des rappels au règlement sur l'interprétation de l'article 45 de la Constitution

par l'autorité compétente, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, des différends susceptibles de surgir sur l'interprétation que nous donnons dans les commissions permanentes, et pas seulement au sein de la commission des lois, de l'article 45 de la Constitution, en croyant juste respecter la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui est plus sévère qu'autrefois.

et la réponse qu'il y apporte va dans la bonne direction. Vous avez mentionné notre collègue député Mansour Kamardine, avec qui j'ai également été en relation ces derniers jours. Il a raison : une meilleure prise en compte des menaces ou des troubles à l'ordre public est nécessaire

en faire l'observation de manière que nous ayons une nouvelle grille de lecture de la recevabilité. C'est simplement une piste parmi d'autres, mais il y a suffisamment de collègues qui se plaignent

une mère et ses quatre enfants, à la suite d'un glissement de terrain, ont trouvé la mort. Voilà aussi les conditions qui sont réservées aux étrangers en situation irrégulière à Mayotte ! J'invite ceux de nos collègues